Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est avec une extrême tristesse et une très vive émotion que nous avons appris

Au nom du Sénat tout entier, je veux saluer le courage et l'abnégation de ces militaires de l'armée de terre- six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef tombés en opération et morts pour la France dans l'essentiel combat contre le terrorisme djihadiste au Sahel. En notre nom à tous, assurer leurs familles de notre profonde compassion et leur présenter nos condoléances les plus attristées. Permettez-moi d'avoir avec vous une une pensée toute particulière pour la famille de notre collègue, dont le fils, jeune lieutenant, figure parmi les disparus. Je viens de Cette nouvelle épreuve est l'une des plus dures qu'ait eue à connaître notre armée depuis le terrible attentat du Drakkar au Liban, en octobre 1983, qui avait D'autres noms vont ainsi, hélas, s'ajouter à ceux des 549 militaires morts pour la France inscrits sur le haut lieu de mémoire nationale, inauguré le 11 novembre dernier en l'honneur de ceux qui ont donné leur vie en opérations extérieures. Je suis certain qu'au moment où nous allons partager ce moment de recueillement vous aurez une pensée pour ces militaires, leurs familles, et plus particulièrement pour celle, chère à notre coeur, de notre collègue, que nous croisons au quotidien dans notre assemblée.

Nous sommes parvenus à l'amendement n° I-394 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 25. L'amendement n° I-394 rectifié, présenté par M. Lurel,

Le présent amendement a pour objet de s'assurer de la cohérence du bénéfice du crédit d'impôt avec le modèle de financement du logement social. Afin de permettre une lecture juste des comptes des organismes de logement social il est nécessaire que le bénéfice du crédit d'impôt s'étale comptablement sur toute la durée de l'opération, comme c'était auparavant le cas avec les dispositifs de défiscalisation. Sans l'adoption de cet amendement, un tel bénéfice continuera d'être comptabilisé sur la seule première année, faussant ainsi les comptes des OLS qui affichent un résultat exceptionnel tandis que ce résultat est largement négatif sur toutes les années suivant le déploiement de l'opération. Cette situation conduit à un défaut de validation des comptes des OLS par les commissaires aux comptes,

Son objectif est de rétablir le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement à l'article 199 C du code général des impôts pour les outre-mer, en le recentrant uniquement sur les opérations de réhabilitation et de rénovation de logements, et en le réservant aux OLS non bailleurs sociaux. Nous prévoyons d'encadrer fortement ce dispositif

La généralisation opérée en loi de finances pour 2019 de l'utilisation du crédit d'impôt prévu à l'article 244 X du CGI n'autorise plus plus les opérations de financement qui permettaient aux personnes à faibles revenus de réaliser un certain nombre de travaux de rénovation et de réhabilitation de leur logement. Les OLS « associatifs

Les propriétaires-occupants qui n'ont pas les moyens de faire les travaux qu'implique l'état d'insalubrité de l'immeuble ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt. Or les besoins sont énormes outre-mer, puisqu'on estime que 13 % des logements y sont insalubres. Dès lors, le rétablissement partiel du dispositif associé à l'article 199 C est indispensable à ces différents acteurs pour maintenir une source de préfinancement et, au-delà, un niveau indispensable de réhabilitation des logements dans les outre-mer. Une telle disposition, qui s'inscrit dans le cadre du nouveau plan logement outre-mer, permettra de poursuivre les opérations impliquées par le plan « Action coeur de ville ».

Nous avions fait des contre-propositions consistant, pour le logement social et la lutte contre l'insalubrité, à mettre en place un prêt à taux zéro de la Caisse des dépôts et consignations,

À cette occasion, des décideurs de tous bords ont alerté le Gouvernement sur la situation particulièrement catastrophique de la Guyane d'un point de vue sanitaire. Ainsi, l'offre de soins en Guyane est marquée par un niveau d'équipement de deux à trois fois inférieur à celui qui est observé dans l'Hexagone, et il existe de forts besoins en matière de périnatalité.

du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est venue simplifier les régimes d'allégements prévus pour les activités économiques réalisées dans les territoires ultramarins. À ce titre, elle a organisé un régime unique, défini par les dispositions de l'article 44 du code général des impôts. qui augmente la quote-part des résultats exonérés pour les entreprises reprises ou créées à compter du 1 janvier 2019, mais en exclut certains secteurs d'activités antérieurement éligibles, parmi lesquels le secteur de la santé. Cette exclusion

de faire mon collègue Maurice Antiste. La loi de finances pour 2019 est venue simplifier les régimes d'allégements prévus pour les activités économiques réalisées dans les territoires ultramarins. À ce titre, elle a organisé un régime unique, qui augmente la quote-part des résultats exonérés pour les entreprises reprises ou créées à compter du 1 janvier 2019, mais en exclut certains secteurs d'activités antérieurement éligibles, parmi lesquels le secteur de la santé. Cette exclusion est venue accentuer les difficultés de recrutement et de maintien des professionnels de santé, en particulier en Guyane et à Mayotte, territoires qui souffrent non seulement d'une pénurie de médecins libéraux, mais également d'une défaillance du service public hospitalier. Très concrètement, alors que l'Hexagone compte environ 437 médecins, généralistes ou spécialistes, pour 100 000 habitants, la Guyane n'en compte que 256 et Mayotte 94. Ces chiffres alarmants, auxquels s'ajoute une forte croissance démographique, laissent craindre une crise sanitaire sans précédent. C'était bien l'objet du débat que nous

l'année 2022, soit quatre ans simplement après Irma. Nous avons pourtant besoin de cet effort. Je ne pourrais pas siéger ici aujourd'hui si je ne défendais pas cet amendement en faveur de mon territoire et de ses acteurs économiques. Nous en avons besoin, monsieur le secrétaire

les dispositions relatives à la réduction d'impôt « s'appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 ou 239 C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 À la lecture de l'article 8 du CGI, on peut constater concrètement qu'à ce jour, lorsque le programme d'investissement est inférieur à 250 000 euros et que l'agrément préalable n'est pas nécessaire, les deux seules formes juridiques de sociétés qui puissent être effectivement utilisées sont la société en nom collectif (SNC) et la société en commandite simple

leur confère une responsabilité solidaire et indéfinie vis-à-vis de la société et un statut de commerçant qui est injustifié, puisqu'ils ne sont, dans les faits, que des associés passifs ne participant pas à l'activité.

ce statut d'associés limite l'engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société. En outre, cette société reste une société de parts sociales, statut plus souple que celui des sociétés par actions, qui sont très réglementées.

Le tissu économique de ces territoires est majoritairement constitué de très petites entreprises. Celles-ci sont peu structurées et mal accompagnées ; un nombre important de prestations juridiques et comptables auxquelles elles ont recours se font dans l'illégalité. Les professionnels du conseil, les consultants, les bureaux d'études techniques et les experts-comptables ayant une activité légale sur ces territoires sont encore trop rares. À titre d'exemple, La Réunion compte actuellement 160 experts-comptables, la Martinique et la Guadeloupe en comptent chacun 80, tandis que l'on en trouve moins de 20 en Guyane et à Mayotte. Si des progrès significatifs ont été réalisés grâce à la baisse des charges sociales, ces efforts ne peuvent à eux seuls combler le retard important de ces territoires par rapport au reste des outre-mer. S'agissant des bureaux d'études, les difficultés rencontrées sont du même ordre. Les secteurs privé et public peinent à faire émerger des projets, à les mener et à assurer leur suivi effectif. Face Face à la sous-consommation des crédits de la mission « Outre-mer », l'État est contraint d'apporter un soutien en ingénierie aux collectivités locales. Il est donc indispensable qu'un appui soit apporté aux bureaux d'études. Enfin, le retour de ces secteurs dans le dispositif des zones franches d'activité nouvelle génération pour la Guyane et Mayotte serait cohérent avec la liste des secteurs prioritaires constituée en matière d'allégements de cotisations sociales.

dans la liste des secteurs bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la zone franche d'activité nouvelle génération. Tel était le

les entreprises industrielles ultramarines sont particulièrement exposées à la double concurrence des pays tiers voisins et de la métropole. C'est pourtant précisément le critère d'exposition à la concurrence externe qui a conduit le législateur, lors de la réforme du régime des exonérations de charges sociales patronales spécifiques à l'outre-mer opérée dans le cadre pour 2019, à intégrer l'ensemble des secteurs industriels dans la liste des secteurs qui peuvent bénéficier du régime majoré. En toute logique, et par parallélisme des formes avec le régime des exonérations de charges sociales patronales, le présent amendement a pour objet d'intégrer les secteurs industriels dans la liste des secteurs bénéficiant des abattements fiscaux majorés des nouvelles Zfang.

du dispositif notamment les activités de réparation et de carénage des bateaux ou encore la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux, tels que les pièces d'accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme,

que les contribuables ultramarins qui font construire ou qui acquièrent un logement neuf bénéficient d'une réduction d'impôt étalée sur dix ans, à la condition qu'ils s'engagent à l'occuper au titre d'habitation principale durant au moins cinq Il est certain que, sans cette aide fiscale, de nombreux contribuables de la classe moyenne auraient été dans l'incapacité financière d'acquérir leur logement. Pour autant, cette réduction d'impôt étant subordonnée à l'affectation du logement au titre de l'habitation principale durant cinq ans,

Dès lors, ils ne peuvent plus bénéficier du crédit d'impôt auquel ils sont éligibles en vertu de cet article. L'amendement a donc pour objet de aux contribuables placés dans l'incapacité de respecter le délai d'affectation à la résidence principale, du fait d'une mobilité professionnelle, de continuer à bénéficier, selon les mêmes règles, de la réduction d'impôt prévue par les textes.

votre proposition, en plus de s'appliquer à un dispositif éteint, inciterait à maintenir des logements inoccupés dès lors qu'elle conditionnerait le bénéfice de la réduction d'impôt à l'absence de mise en location du bien. Je ne pense pas que votre objectif soit d'empêcher la location ces biens. Je maintiens

est ainsi libellé : La parole est à M. Michel Magras. Cet amendement vise à introduire un mécanisme de réduction d'impôt en remplacement de la déduction du résultat imposable des investissements ou souscriptions au capital dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. De fait, la baisse progressive du taux d'imposition sur les sociétés réduit, pour les entreprises fiscalement domiciliées en métropole, l'attractivité fiscale de ces investissements ou souscriptions dans ces collectivités et en Nouvelle-Calédonie. Pour maintenir un nécessaire apport en capital dans ces territoires, il est proposé une réduction d'impôt à à taux fixe à hauteur de 35 %, identique au taux du crédit d'impôt applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés par l'article 244 W du code général des impôts pour les investissements productifs qu'elles réalisent dans les

il n'est pas établi que la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés affectera le flux des investissements outre-mer. Nous ne disposons d'aucune donnée pouvant corroborer cette hypothèse. Surtout, la mesure proposée entraînerait un effet d'aubaine pour des investisseurs personnes morales soumis à l'impôt sur les sociétés en métropole, qui bénéficieraient à la fois de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés et d'un avantage fiscal au moins égal à celui qui est actuellement octroyé. Il ne nous paraît pas opportun de modifier l'équilibre actuel. L'engagement a été pris

-, dans celui des arts plastiques ou dans celui de la littérature. De façon générale, il ressort que les outre-mer, notamment la Martinique, concentrent de nombreux talents,

le déplacement d'un objet d'art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en oeuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens. Cet amendement Cet amendement a donc pour objet d'alléger la fiscalité applicable aux biens culturels dans les départements et collectivités d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, en les exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nos nombreuses tentatives de parvenir à l'égalité, voire à l'équité, butent sur d'incompréhensibles refus.

n'arrivent pas à vivre du fruit de leur imagination ou de leur création. À l'heure où l'on remet en cause le soutien au mécénat,

de 323 millions d'euros par rapport à 2019. Cela s'explique par plusieurs évolutions : d'abord, la progression des compensations d'exonérations de fiscalité locale, 123 millions d'euros, ainsi que celle du Fonds de compensation pour la TVA

Certes, une telle augmentation globale est incontestablement positive, mais la réduction des variables d'ajustement pose problème. En effet, dans une moindre mesure par rapport aux années précédentes, les dotations de compensation sont minorées de 120 millions d'euros, afin de maîtriser la hausse tendancielle des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales par rapport au niveau des crédits fixé en loi de finances initiale pour 2019. Il s'agit donc d'une nouvelle baisse intégrant pour la première fois le versement transport qui sera amputé quasiment de moitié. De même, les régions devront renoncer à 55 millions d'euros de dotations, dont 35 millions d'euros au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Tels sont, mes chers collègues, les quelques points très négatifs que nous souhaitons mettre en exergue préalablement à l'examen de l'article.

pour 2020, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont estimés à 40,9 milliards d'euros, dont une grande part, 26,8

et d'investissements. Le prélèvement sur recette au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est de 2,4 milliards d'euros. La dotation de compensation

fondamentalement. Premièrement, l'affaiblissement régulier depuis des années des dotations financières aux communes les empêche de mettre en oeuvre les programmes pour lesquels ils ont été élus afin de répondre aux aspirations de la population.

la collectivité. Certains ne se versent même pas d'indemnité ! Une telle réévaluation répondait à une réelle nécessité de valorisation des fonctions remplies par les maires et adjoints de petites communes. que, comme beaucoup d'élus nous le disent sur le terrain, si l'augmentation du plafond d'indemnisation ne s'accompagne pas de moyens supplémentaires, cela ne sert strictement à rien !

seulement. Cela nous paraît néanmoins insuffisant au regard des besoins. Faisons un petit calcul : 28 millions d'euros, cela fait très exactement 1 305,23 euros de plus par an par commune, soit 108,76 euros de plus par mois pour les indemnités du maire et des adjoints.

à la ruralité. Ces 65 millions d'euros de plus, soit 3 030 euros de plus par commune, équivalent à 252,50 euros supplémentaires par mois

la rétrocession aux communes guyanaises de la part du produit de l'octroi de mer prélevée au profit de la collectivité territoriale de Guyane a été compensée par un prélèvement sur les recettes de l'État. pour 2020 prévoyait de prolonger le versement de la compensation de l'octroi de mer à la collectivité territoriale de Guyane à hauteur du montant versé en 2019, soit 27 millions d'euros, sous la forme d'une dotation en contrepartie de la mise en oeuvre d'une maîtrise de ses dépenses. La préparation d'une convention d'objectifs de performance entre l'État et la collectivité territoriale de Guyane est en cours et devrait aboutir à la signature d'un accord de méthode dans les prochains jours. Eu égard au sérieux des travaux engagés à l'échelon local, il est proposé de rétablir le prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane, à un montant évalué à 27 millions d'euros pour 2020. Cet amendement vise donc à tenir compte dans le total des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales du rétablissement en PSR

à la question des parcs nationaux et des parcs marins -et, d'autre part, à traduire l'engagement pris par le Premier ministre devant le Congrès des maires, à hauteur de 28 millions d'euros. Cela correspond à la prise en charge qui serait rendue nécessaire

La mise en place de communes nouvelles laisse inchangé le nombre d'élus locaux jusqu'à la fin du mandat. Cela a souvent pour conséquence de diminuer fortement le nombre de communes éligibles, alors que les charges afférentes à chaque commune demeurent.

je pense à la couverture numérique, à l'enfouissement des réseaux électriques, à la conversion du parc électrique en leds pour réaliser des économies d'énergie -et sur les réseaux humides. L'adoption de cet amendement

Il intègre ainsi les besoins d'entretien urgents et importants identifiés à la fois sur les réseaux humides et sur les réseaux secs, tels que la couverture numérique, l'enfouissement des réseaux électriques ou la conversion du parc électrique en leds pour réaliser des économies d'énergie.

pourtant une infrastructure, mais utilisée sous forme de prestation de services. Je propose de l'inclure dans ce qui relève du remboursement au titre du FCTVA,

En 2019, le parc automobile des collectivités territoriales représente 150 000 véhicules, dont 74 % de véhicules diesel, 18 % de véhicules à essence et seulement 8 % de véhicules électriques. Comme mes collègues, j'estime

ont été appelés à participer à l'effort budgétaire en raison du contexte économique et conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Cette contribution est bien évidemment compréhensible, mais elle ne doit en aucun cas être disproportionnée ni aboutir à remettre en cause l'existence même de ces structures appelées à l'effort de redressement des comptes publics. publics. En effet, une diminution des ressources de ces organismes à hauteur de 124 millions d'euros serait excessive, ne manquerait pas de les déstabiliser et les empêcherait de réaliser

prélevés sur les assurances habitation pour alimenter ce fonds. Celui-ci appartient donc aux assurés, qui doivent en avoir le juste retour lorsqu'ils subissent des catastrophes naturelles.

Depuis 2012, on trouve parmi les taxes affectées plafonnées, dont il est ici question, les taxes finançant les centres techniques industriels, Ces taxes sont acquittées par les industriels des différentes filières et ces sommes sont consacrées à l'activité des CTI, qui sont chargés de faire ruisseler l'innovation jusqu'aux plus petites entreprises et de mettre en place des projets de R&D, ou « politiques de transfert sont implantés dans les territoires, sur environ 50 sites, auprès des PME. Voilà sept ans que ces taxes sont plafonnées. Concrètement, l'État confisque chaque année 14 millions d'euros destinés à l'action industrielle pour les reverser au budget général. Nous n'avons cessé de déplorer ce plafonnement et ses conséquences sur la modernisation de l'industrie, y compris l'année dernière, quand le Gouvernement décidait de baisser une nouvelle fois les plafonds.

affectées aux CTI. En l'espèce, le Gouvernement entend déplafonner quatre nouvelles taxes. Nous devons nous en féliciter, mais il faut aller au bout des choses. Six CTI, dont ceux du secteur du bois, des papiers et cartons ou de la bijouterie, se verront encore cette année privés de ressources qui leur reviennent de droit. Malheureusement, les règles de recevabilité des amendements ne nous permettent pas de demander le déplafonnement des taxes restantes. Monsieur le secrétaire d'État, je m'adresse donc à vous : vous engagez-vous, devant le Sénat, à déplafonner dès maintenant les taxes affectées à tous les CTI, afin de ne pas prendre davantage de retard dans l'effort d'innovation nécessaire à nos PME, TPE et ETI ?

secrétaire d'État. Le droit de timbre étant géré conjointement avec les redevances cynégétiques, il était cohérent de l'affecter également aux agences de l'eau, ce qui a été fait lors des débats à l'Assemblée nationale. Il reste maintenant à assurer la neutralité de la mesure aux opérateurs de la biodiversité.

lors que les centres signent un contrat avec l'État comprenant des objectifs de restructuration et de modernisation. L'excellent rapport de Mme la députée Anne-Laure Cattelot nous a permis de fixer une méthodologie. Depuis l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale,

l'amendement n° I-966 rectifié. La loi de finances pour 2016 a créé deux recettes extrabudgétaires de nature fiscale qui abondent les moyens alloués à l'aide juridictionnelle, pour un montant annuel de 83 millions d'euros. Il s'agit, d'une part, d'une taxe sur les assurances de protection juridique, à hauteur de 45 millions d'euros, d'autre part, d'un prélèvement forfaitaire sur le produit d'une partie des amendes pénales, à hauteur de 38 millions Le produit de ces recettes extrabudgétaires pour l'aide juridique est géré par le Conseil national des barreaux, qui représente la profession d'avocat, puis réparti entre les barreaux pour la rémunération des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle.

Cet amendement vise à maintenir le dispositif d'affectation existant, qui a montré son efficacité, notamment grâce à des rapports de gestion précis et réguliers de consommation faits au ministère de la justice. Il est nécessaire que soit conservé le lien entre l'assurance de protection juridique et l'accès au droit. Dans l'attente de l'évolution nécessaire de l'assurance de protection juridique- extension à de nouveaux domaines, meilleure information des assurés sur leurs garanties -, la taxation des contrats pour financer l'aide juridictionnelle conserve toute sa cohérence. Le secteur de l'assurance de protection juridique est depuis plusieurs années le plus rentable de l'activité des compagnies d'assurance.

Depuis plus de deux ans, nous attendons le débat parlementaire sur un projet de loi réformant en profondeur l'audiovisuel public, mais je ne peux m'empêcher de me demander de quoi nous discuterons réellement. En effet, depuis les fuites sur le rapport CAP 22, on sent que toutes les décisions ont déjà été prises et mises en application.

dans un contexte de construction des dotations de l'État en direction du groupe audiovisuel public. Un débat législatif devrait avoir lieu sur les sources de financement du groupe, mais le débat budgétaire est la seule opportunité de discuter du financement.

Par souci de cohérence budgétaire, il est proposé de revenir au taux initial de 0,9 % pour en réduire le poids. Créée par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision pour compenser la baisse des ressources résultant de la suppression partielle de la publicité sur les antennes de France Télévisions, la taxe due par tout opérateur de communications électroniques (TOCE) a été affectée de manière résiduelle au groupe public jusqu'en 2018. Initialement fixé à 0,9 % du montant hors TVA des abonnements et sommes acquittés par les usagers aux opérateurs, son taux a été majoré de 44 % par la loi de finances pour 2016, à hauteur de 1,3 %, dans le but d'affecter des ressources supplémentaires à France Télévisions. Ce dispositif, qui ampute fortement les capacités d'investissement des opérateurs-

du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision pour compenser la baisse des ressources résultant de la suppression partielle de la publicité sur les antennes de France Télévisions, la taxe due par tout opérateur de communications électroniques, dite TOCE ou taxe Copé, lui était affectée de manière résiduelle jusqu'en 2018. Il n'y a rien d'incohérent Initialement fixée à 0,9 % du montant hors TVA des abonnements et sommes acquittés par les usagers aux opérateurs, son taux a été majoré de 44 % par la loi de finances pour 2016, à hauteur de 1,3 %, dans le but d'affecter des ressources supplémentaires à France Télévisions. Ce dispositif, qui ampute fortement les capacités d'investissement des opérateurs, n'entretient donc plus aucun lien avec sa raison d'être, le financement de l'audiovisuel public. La loi de finances pour 2019 ayant supprimé la part de la taxe affectée à France Télévisions,

sans créer de nouveaux péages pour les usagers ou les transporteurs. Ensuite, nous devons corriger une incohérence dans le dispositif global. En effet, chaque année, le montant des tarifs de péage des sociétés d'autoroutes augmente d'au moins 70 % du montant de l'inflation, alors que, dans le même temps, le taux de la taxe d'aménagement du territoire est gelé. gelé. L'indexation que nous proposons ne remet pas en cause le modèle économique des sociétés d'autoroutes. Avec l'indexation, le montant supplémentaire de la TAT sera de l'ordre de 5 millions d'euros par an, sur un chiffre d'affaires global des sociétés d'autoroutes représentant plus de 10 milliards d'euros. Nous pouvons donc considérer que ce montant est relativement marginal.

mes chers collègues, qu'il y a un an commençait le grand épisode des « gilets jaunes » lesquels en avaient largement contre les sociétés d'autoroutes. Il faut se souvenir des réclamations

Il vise à supprimer les sous-plafonds du fonds Barnier qui ne fonctionnent pas vraiment, afin de donner davantage de souplesse à la gestion de ce fonds

qui constitue une aggravation des charges publiques au sens de l'article 40 de la Constitution- c'est une jurisprudence constante et ancienne de la commission.

droits et obligations au bénéfice des nouveaux opérateurs de compétences, sous réserve que ces derniers interviennent avant le 31 décembre 2019. Or la loi et ses textes d'application ont réformé en profondeur le financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle, ce qui a entraîné dans les faits un glissement du calendrier initialement envisagé. Les OPCA ne seront pas en mesure de finaliser la procédure de transfert des biens immobiliers vers les nouveaux OPCO avant le 31 décembre prochain et ne pourront donc pas bénéficier de l'exonération de droits de mutation et de la contribution visée à l'article 879 du code général des impôts. En conséquence, le présent amendement vise à modifier l'échéance initialement fixée par la loi, en retenant la date du 30 juin 2020 pour réaliser l'ensemble des opérations de transfert, tout en bénéficiant des exonérations fiscales initialement prévues.

pour établir un diagnostic sur la gestion et l'action des fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées. L'objectif est de proposer des pistes de réforme pour améliorer l'efficience et la transparence de leur gestion dans le mouvement engagé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. L'enjeu porte sur environ 330 millions d'euros de collecte en 2017 pour 3,2 millions de travailleurs indépendants, soit 11 % de la population active. Parallèlement, la loi en question et l'ordonnance du 21 août 2019 ont confié à France compétences le soin d'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle. Dans ces conditions, il paraît logique que les excédents financiers constatés dans l'une des structures visées par cet amendement soient directement versés à France compétences, afin que cette institution soit en mesure d'assurer ses obligations légales en matière de financement de la formation professionnelle et de l'alternance.

l'audiovisuel public devrait voir sa dotation publique baisser au total de 190 millions d'euros entre 2019 et 2022, dont 161 millions seront imputables sur la seule dotation de France Télévisions et 20 millions sur celle de Radio France. Il reste donc encore 155 millions d'euros d'économies à réaliser sur les trois prochains exercices budgétaires. En plus d'être hypocrite, cette mesure est manifestement idéologique, puisque son unique objet est d'asphyxier économiquement l'audiovisuel public.

le président Sarkozy avait décidé d'interdire aux chaînes publiques de commercialiser des espaces publicitaires en soirée. En 2018, le Gouvernement a décidé d'interdire la publicité dans les programmes pour la jeunesse de France Télévisions, ce qui correspond à une perte de recettes de 17 millions d'euros. Enfin, en cette rentrée, le ministre de la culture a fermé la porte

l'audiovisuel public a déjà subi des coupes budgétaires et réalisé des économies depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il arrive à un point de non-retour extrêmement préoccupant.

régler les problèmes de pouvoir d'achat des Français ; en revanche, elle sera extrêmement douloureuse pour l'audiovisuel public. Ceux qui écoutent les radios du service public savent que les personnels sont en grève depuis hier. Nous les Nous les avons rencontrés : ils nous ont décrit la réalité de leurs missions dans le contexte budgétaire qui est le leur, avec à la fois un gouvernement qui demande des économies et une direction qui applique les mesures plutôt avec zèle, à mon avis. mon avis. Dans un contexte où la parole publique est aussi contestée et sujette à caution, nous avons besoin d'un audiovisuel public fort, pluraliste,

d'autres pays où la décentralisation est plus aboutie, des médias locaux avec des participations plus fortes et des débats mieux organisés.

et les biens mal acquis, qui constituent un véritable pillage des pays les plus pauvres de la planète par des personnes malhonnêtes, qui accumulent des biens en France, à Paris, sur la Côte d'Azur et ailleurs.

Jean-Pierre Sueur a rappelé, à juste titre, la position unanime du Sénat sur la restitution des biens mal acquis,

entre les auteurs du texte et le Gouvernement, non pas sur l'objectif, mais sur les modalités. Nous avions notamment échangé ensemble sur la nécessité de modifier la loi organique fixant les compétences de l'Agrasc pour pouvoir permettre l'affectation particulière.

fonds et un conseil pour gérer ce fonds, de telle manière que les biens volés reviennent aux populations qui ont été spoliées.

En effet, après des années d'efforts- en particulier du gouvernement précédent, il faut le saluer, mais d'autres aussi -, la sécurité sociale est revenue globalement à l'équilibre financier.

même que nous savons les Français inquiets pour leur protection sociale et que le Gouvernement reconnaît lui-même l'ampleur des besoins pour financer les mesures en faveur du grand âge,